Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au cours des dernières semaines, les outre-mer ont été confrontés à la pire crise sanitaire que notre pays ait connue depuis le début de l'épidémie de covid-19. Ce constat, c'est le ministre des outre-mer lui-même, Sébastien Lecornu, qui l'a dressé le 9 septembre dernier au Sénat lors du débat sur le projet de loi relatif à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer. Le rapporteur de la commission des lois, notre collègue Philippe Bas, qui est également membre de la délégation sénatoriale aux outre-mer, a eu des mots très forts pour évoquer cette situation : « Aujourd'hui, nous sommes tous Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Polynésiens ... Nous sommes tous ultramarins. Nous avons tous une pensée pour nos compatriotes qui sont si nombreux dans le deuil, la souffrance de la maladie, l'angoisse, quand on voit l'épidémie se répandre à une vitesse dont nous n'avions jamais fait l'expérience.

C'est ce contexte inédit dans les outre-mer, avec des pics jamais atteints auparavant, que nous devons avoir à l'esprit, alors que s'ouvre la présente session parlementaire 2021-2022 et que l'occasion nous est offerte de rappeler le lourd tribut que notre pays, et les outre-mer en particulier, a payé et continue de payer à cette pandémie.

en séance publique sur la politique du logement -pour nous consacrer entièrement à la situation sanitaire dans les outre-mer. Je tiens à remercier les rapporteurs Victorin Lurel, Micheline Jacques et Guillaume Gontard, qui ont d'emblée soutenu cette démarche et ont permis qu'un débat s'organise en priorité sur ce sujet, afin de prendre la mesure de la situation d'urgence sanitaire, encore très prégnante dans nos territoires. Même si cette situation évolue, et on a vu au cours de ces derniers temps à quel point l'évolution pouvait être fulgurante, un tel phénomène interpelle l'ensemble de la représentation nationale. Les taux d'incidence, le nombre de victimes, la « priorisation » durant certaines phases aiguës, la mobilisation et le dévouement extraordinaires des équipes de soignants, que nous saluons, le recours à la réserve sanitaire ... tous ces faits récents nous conduisent à nous interroger sur la gestion de la crise, sur son efficacité et sur les leçons à en tirer pour chacun de nos territoires. Par ailleurs, comme vous le savez, le président Gérard Larcher a aussi souhaité que la mission commune d'information du Sénat sur les effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restrictions d'activités- la mission est présidée par notre collègue Bernard Jomier et ses rapporteurs sont Jean-Michel Arnaud et Roger Karoutchi -se saisisse de la situation spécifique des territoires ultramarins pour en examiner les conséquences tant sanitaires qu'économiques et sociales. Elle va ainsi se pencher sur les causes de la dernière vague épidémique et dégager des préconisations. Les travaux de la mission ont démarré la semaine dernière, avec une table ronde

La mission commune va organiser notamment des tables rondes géographiques permettant de mieux appréhender la situation propre à chaque territoire. Je tiens à saluer la démarche dans laquelle la mission a choisi de s'inscrire. Celle-ci est de nature à permettre une analyse approfondie et territorialisée. En effet, les situations sont très contrastées. Il existe des territoires qui, jusqu'à présent, ont été plus ou moins épargnés et qui ont pu prévenir la propagation du virus, alors que d'autres sont très durement frappés. Naturellement, on ne fera pas l'économie du débat sur le taux de vaccination, sujet sur lequel beaucoup a déjà été dit, mais il est aussi important, comme l'ont souligné nos collègues Victoire Jasmin, Jocelyne Guidez ou Victorin Lurel lors de la première audition, d'appréhender les aspects information et communication sur le sujet. Ce n'est pas un hasard si, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, les parlementaires souhaitent que l'on approfondisse les modalités d'anticipation et de gestion de la crise. Comme l'a indiqué l'une des personnes auditionnées le 28 septembre dernier : « Il faut utiliser les prochaines semaines pour se préparer nationalement et localement à une possible cinquième vague, qui, hélas, adviendra probablement. » La crise sanitaire appelle à faire preuve de responsabilité. Hôpitaux saturés, lits de réanimations débordés, appels à la réserve sanitaire, évacuations sanitaires spectaculaires, prorogations de l'état d'urgence ... la dégradation soudaine de la situation sanitaire dans certains territoires s'est traduite par des images-chocs et des bilans dramatiques. La pandémie a éclairé sous une lumière crue la réalité de l'offre de soins dans les outre-mer. C'est cette réalité qu'il convient aussi de regarder en face. Nos inquiétudes sont également sont également d'ordre économique. Notre délégation s'est saisie très tôt, dès le mois d'avril 2020, des conséquences de la pandémie de covid-19 sur les économies ultramarines, déjà fragilisées. Avec mes collègues Viviane Artigalas et Nassimah Dindar, nous avons dressé un premier état des lieux et produit une soixantaine de recommandations sur l'urgence économique outre-mer. La mission pourra s'appuyer sur ces travaux, ainsi que sur ceux du Conseil économique, social et environnemental et sur ceux des chambres de commerce et d'industrie des outre-mer, car ils restent d'actualité. Au fil de nos auditions, la délégation s'était non seulement intéressée aux mesures d'urgence mises en place pour sauvegarder le tissu économique dans les outre-mer, mais elle avait aussi identifié des secteurs clés- tourisme, secteur aérien, BTP -, à soutenir après la quasi-mise à l'arrêt des activités. Elle avait également alerté sur la situation financière dégradée des collectivités locales, qui méritent aussi un accompagnement adapté. Nos collègues nous ont d'ores et déjà alertés sur la hausse générale des prix des matières premières, du coût du fret, du prix de l'énergie et, au-delà, de nombreux intrants.

Nous devons absolument y apporter des réponses si nous ne voulons pas continuer à subir les vagues épidémiques et leurs conséquences humaines, économiques et sociales ravageuses.

Quels efforts budgétaires et quels investissements pouvez-vous annoncer pour les prochains mois ? Compte tenu des disparités persistantes constatées selon les territoires, avec actuellement une sorte de « plateau vaccinal », comment allez-vous renforcer la pédagogie autour de la vaccination ? Comptez-vous par ailleurs renforcer le rôle des instances de dialogue et de concertation, comme les conseils territoriaux de santé ? Quels moyens supplémentaires seront mis en oeuvre pour former et recruter davantage de personnels, mieux les équiper et les rétribuer ? Comment comptez-vous améliorer les possibilités d'évacuation sanitaire, comme l'élément militaire de réanimation (EMR), et adapter ces moyens à l'isolement et au caractère insulaire, voire archipélagique ? Voilà quelques-unes des nombreuses questions que nous voulions vous soumettre, monsieur le secrétaire d'État. Je laisserai bien entendu mes collègues, que je remercie chaleureusement de leur présence, les compléter. Je ne doute pas que le débat sera riche. Nous attendons des réponses précises

En un peu plus d'un an et demi de crise sanitaire, la situation dans les différents territoires d'outre-mer a fortement varié, avec des trajectoires propres à chacun d'entre eux.

les systèmes de soins et les organisations publiques. Vous le savez, les difficultés tiennent en grande partie à la contagiosité accrue du variant delta, mais également à une faible couverture vaccinale, ainsi qu'à des facteurs saisonniers ou structurels face auxquels nous devons sans cesse adapter notre stratégie. La concomitance et l'intensité des vagues épidémiques ont justifié l'adoption de mesures de freinage fortes

Pour alléger la pression hospitalière, des renforts ont été mobilisés, avec notamment l'arrivée de cinquante personnes samedi dernier. Cette aide permet d'ouvrir de nouveaux lits de réanimation et de compenser une partie des arrêts maladie des personnels soignants.

des soignants, qui sont surmobilisés. Là aussi, renforts et évacuations se sont multipliés. Les équipes sanitaires travaillent quotidiennement à la définition du besoin précis pour que les missions puissent être menées à bien. Ailleurs, la situation s'est améliorée, y compris très récemment. Dans les Antilles, la situation, tant épidémiologique qu'hospitalière, est meilleure. Les indicateurs continuent ainsi d'aller dans le bon sens en Guadeloupe et en Martinique, avec des taux d'incidence en forte baisse. En Guadeloupe, le déconfinement a débuté le 22 septembre selon un plan en trois phases, mais la vigilance doit évidemment rester de mise. À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la situation est également de plus en plus favorable. Il en va de même à la Réunion, où la situation sanitaire continue aussi de s'améliorer, avec une poursuite du ralentissement de la circulation virale et une diminution du nombre d'hospitalisations, d'admissions en de décès. En Polynésie française, la tendance générale est également à la baisse des indicateurs, permettant d'envisager une levée progressive du couvre-feu. À Mayotte, les indicateurs épidémiologiques sont en diminution depuis plusieurs semaines, mais la prudence doit rester de mise. Je le répète après vous, monsieur le président, nous devons rester vigilants. Là où les données montrent une amélioration, elles montrent aussi parfois, non pas un relâchement, mais une moindre mobilisation, notamment autour des dépistages. La communication, l'information, la pédagogie et la sensibilisation doivent se poursuivre auprès des populations, des relais d'opinion et des relais communautaires pour rappeler les gestes barrières et l'importance de la vaccination. Les efforts en matière de campagne vaccinale doivent être poursuivis. La vaccination, c'est justement ce qui permet et permettra, de plus en plus, d'améliorer la situation hospitalière. Débutée très tôt, puisque les premières doses sont arrivées dès janvier dans de nombreux territoires, la campagne vaccinale est montée en puissance progressivement, mais ne permet pas encore aujourd'hui de produire les effets attendus, du fait, vous le savez, de réticences extrêmement fortes. La vaccination atteint un niveau satisfaisant à Saint-Pierre-et-Miquelon et s'en rapproche à la Réunion et en Polynésie, même si elle doit bien sûr être encore encouragée. La dynamique est également plutôt positive en Nouvelle-Calédonie, mais les efforts doivent se maintenir. Trop de territoires restent cependant en retard dans cette campagne de vaccination. En Martinique, la couverture vaccinale demeure insuffisante, et laisse craindre un retour à des niveaux élevés de circulation de virus si les mesures de freinage étaient levées trop rapidement. Même chose en Guadeloupe, où la rentrée scolaire a fait l'objet d'une vigilance renforcée. Si les taux de vaccination n'augmentent pas, une nouvelle vague n'est malheureusement pas à exclure. La Guyane se distingue malheureusement par une vaccination très limitée en population générale, mais aussi chez les soignants. Enjeu peut-être sous-estimé au départ, la lutte contre les fausses informations a fait l'objet d'une mobilisation complète de l'ensemble des acteurs concernés. C'est un effort collectif indispensable pour renforcer l'adhésion de nos concitoyens aux mesures nécessaires à la lutte contre l'épidémie. Je parlais de la Guyane à l'instant. Les opérations « d'aller vers » y sont massives depuis des mois ; la promotion vaccinale y est adaptée aux différentes langues du pays, et est assurée par des professionnels et des associations de terrain, que je remercie pour leur engagement. Pourtant, les chiffres restent insatisfaisants. Les enquêtes sur l'hésitation vaccinale conduites régulièrement laissent craindre une véritable épidémie de fausses informations, et une instrumentalisation des inquiétudes relatives au vaccin. Il nous faut compter sur l'engagement de tous pour dépasser cette situation. À Mayotte, l'agence régionale de santé (ARS) a déployé une communication extrêmement large, diversifiée, traduite en shimaoré, par exemple,

avec les élus locaux, sur le terrain, pour déconstruire les messages fantaisistes et alarmistes que certains se plaisent à diffuser. Je tiens à saluer la mobilisation d'un grand nombre d'entre vous et j'invite tous les élus à rejoindre ce mouvement, en responsabilité. Depuis le début, nous affrontons ensemble cette crise sanitaire. Par-delà les différends politiques et les critiques liées aux méthodes, aux organisations ou aux temporalités- nous y reviendrons -, je pense que nous devons toujours nous retrouver lorsqu'il s'agit de garantir la sécurité et la bonne santé de nos compatriotes ultramarins. Évidemment, la vaccination n'est pas l'unique sujet à l'ordre du jour. Parfois confrontés à des situations difficiles, devant s'accommoder de mesures d'ordre public strictes mais nécessaires, les citoyens de l'ensemble des territoires d'outre-mer ont fait preuve d'une résilience et d'une solidarité

Des renforts continuent ainsi à être mobilisés autant que de besoin pour appuyer les territoires en difficulté. Au plus fort de la crise, et encore aujourd'hui, le Gouvernement a donc mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour apporter la réponse adaptée aux enjeux précis des différents territoires d'outre-mer, avec leurs spécificités. d'outre-mer, avec leurs spécificités. Les énergies ont été mobilisées, les organisations utiles ont été trouvées, et les défis logistiques ont été relevés. À nous, collectivement, de garantir que cela continuera à l'avenir, bien au-delà de la crise sanitaire. C'était le sens de vos propos, monsieur le président, et c'est l'engagement du Ségur de la santé, dont les premiers effets se font sentir, avec force, dans les territoires d'outre-mer. Ensemble, le Gouvernement, les parlementaires, les élus et autorités locales continueront ce travail partenarial qui a fait ses preuves, permettant qu'à aucun moment de la crise le moindre territoire de la République ne soit délaissé, abandonné ou mis de côté. Les outre-mer, dans toute leur diversité, leurs forces respectives, leurs préoccupations spécifiques, ont traversé et continuent de traverser cette crise sanitaire, certes en lui payant un lourd tribut, tribut, mais en pouvant compter, dès la première seconde et jusqu'à la dernière, sur la solidarité de la Nation tout entière. Que cela soit pour moi l'occasion de remercier une fois encore l'ensemble des équipes du secteur sanitaire et social, au sein de l'Hexagone comme dans les outre-mer. Je me tiens désormais à votre disposition pour

et sont des victimes directes de l'épidémie de covid-19, alors même que le virus est généralement sans gravité pour eux. Voilà plus d'un an et demi que nos enfants, nos adolescents se trouvent régulièrement, et pour de longues périodes, éloignés de leurs établissements scolaires. En 2019, avant cette crise, les taux d'illettrisme dans nos territoires étaient déjà alarmants : 35 % des jeunes faisant leur Journée défense et citoyenneté avaient des difficultés de lecture en Martinique, 30 % en Guadeloupe et 50 % à Saint-Martin, quand la moyenne nationale se situait à 11,8 % mois qui viennent de s'écouler auront sans doute, malheureusement, aggravé cette situation dramatique. Vous savez, monsieur le secrétaire d'État, que l'enseignement à distance pose problème, chez nous peut-être encore plus qu'ailleurs, tant les inégalités sociales sont marquées. Tous nos enfants n'ont pas forcément accès à un ordinateur ou à Internet, et tous nos parents ne sont pas en mesure d'aider dans le travail scolaire ... Deux enfants sur trois vivent dans des familles monoparentales, dont les mères ne sont pas toujours accompagnées pour faire face à cette situation qui perdure. Il était certes nécessaire de repousser la rentrée aux Antilles, et je ne le discute pas, mais le retour à l'école doit être une priorité absolue, de même que la mise en place urgente de mesures ambitieuses de soutien pour que les enfants qui ont souffert de la situation puissent rattraper leur retard. Que faites-vous, que comptez-vous faire pour que les chances futures de nos enfants ne soient pas durablement compromises par la période que nous venons de traverser ?

niveau national, les données dont dispose aujourd'hui le ministère de l'éducation nationale montrent que les retards pris avec la crise sont en passe d'être rattrapés et compensés.

sommes fiers de cet engagement des équipes éducatives. Nous ajoutons une volonté forte de poursuivre au bénéfice des élèves les transformations qui sont engagées depuis 2017, en dépit des aléas de la crise sanitaire. Cela passe par l'élévation du niveau général et l'égalité des chances, avec la volonté d'assurer partout

Nous l'avions rappelé unanimement, cette situation de catastrophe sanitaire est la résultante de nos vulnérabilités structurelles et des faibles taux de vaccination. Sur ce dernier point, les causes sont multiples et complexes, dans des territoires où la méfiance envers les institutions de l'État est nourrie chaque jour par une désinformation accrue, engendrée par des diplômés des réseaux sociaux plutôt que par des facultés de médecine. À cela peut s'ajouter une communication des autorités sanitaires jugée parfois trop généraliste dans certains territoires. Depuis, nous avons voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer jusqu'au 15 novembre 2021. Un mois après ce dixième texte d'urgence, où en sommes-nous ?

comment pourrons-nous affronter une prochaine vague avec des systèmes de santé si fragiles ? Que prévoit le Gouvernement pour permettre à nos territoires structurellement en retard de se doter d'un système de santé plus résilient et robuste ? Avant de conclure mon propos, je tiens à saluer le courage de nos collègues Georges Patient, Teva Rohfritsch ou encore Catherine Conconne, qui ont adopté une ligne claire face aux colporteurs d'inepties et de contrevérités. Le mensonge prend souvent l'ascenseur, tandis que la vérité passe par l'escalier. Ne craignons pas d'emprunter collectivement cet escalier ! La parole est à M. le secrétaire

l'adoption de mesures de freinage fortes et précoces. Leur maintien dans la durée est parfois nécessaire, y compris là où la circulation virale baisse, pour éviter une résurgence. Cette stratégie est exigeante,

évidemment compter jusqu'au bout sur le soutien du Gouvernement, même s'il n'y a malheureusement pas de recette miracle. Il faut continuer à mobiliser la solidarité nationale, à envoyer des renforts tant que cela est nécessaire et à maintenir en tension des dispositifs qui ont fait leurs preuves, si besoin au moyen d'actions de communication. À Mayotte, les enjeux sont clairs : si les indicateurs épidémiologiques sont en diminution depuis plusieurs semaines, le territoire demeure particulièrement fragile et vulnérable, la principale raison étant la faible couverture vaccinale. En effet, seuls 44 % de la population globale à Mayotte disposent d'au moins une dose de vaccin.

Les chiffres sont alarmants, du fait notamment de la contagiosité accrue du variant delta. Les hôpitaux doivent faire face à un afflux massif de malades : les services de réanimation sont saturés, les urgences débordées En Nouvelle-Calédonie, où la vaccination a pourtant démarré en janvier, 32 % seulement de la population disposent d'un schéma vaccinal complet. ce faible taux se greffent les modes de vie communautaires océaniens et les multiples comorbidités qui frappent les Calédoniens, offrant un terrain propice au désastre sanitaire en cours. La barre des 100 morts a été franchie la semaine dernière. La situation sanitaire est aussi sombre en Guyane, où le taux d'incidence grimpe en flèche, alors qu'une large partie de la population reste, elle aussi, rétive, voire hostile au vaccin. Les chiffres le démontrent : moins de 25 % des Guyanais sont totalement vaccinés. En conséquence, l'épidémie ne faiblit pas, et le nombre de décès atteint des niveaux inédits. Est-il acceptable de voir des soignants « anti-vaccins » manifester devant un hôpital ? Monsieur le secrétaire d'État, cette épidémie est devenue, dans les outre-mer, une épidémie des « non-vaccinés Face à ce drame, il y a urgence à agir, et la solution, nous le savons tous maintenant, c'est la vaccination. Aussi, envisagez-vous de rendre obligatoire la vaccination dans les territoires ultramarins les plus touchés

toujours par une forte tension. Nous espérons toutefois qu'un plateau a été atteint. Pour traverser cette période difficile, 291 professionnels de santé ont été envoyés sur place depuis l'Hexagone. Plusieurs tonnes de matériel et de produits de santé ont également été envoyées. La coopération entre la Nouvelle-Calédonie,

mais elle est actuellement en pleine quatrième vague épidémique, avec une forte tension hospitalière et une situation particulièrement fragile qui nécessitera probablement des mesures supplémentaires.

pour freiner, et peut-être un jour arrêter l'épidémie. Elle réduit considérablement les risques de formes graves de la covid-19 et, plus important encore, le nombre de décès. Les études scientifiques l'ont montré. La « vie réelle » l'a montré également : les territoires les plus vaccinés sont aujourd'hui ceux où l'épidémie est la moins virulente et les décès les moins nombreux. La vaccination est efficace, ouverte à tous, prise en charge à 100 %. Mais alors que notre pays a la chance de disposer de vaccins, force est de constater que la couverture vaccinale du territoire est très hétérogène, les territoires ultramarins étant loin derrière la moyenne nationale. Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, Guyane : dans aucun de ces territoires, le taux de personnes avec au moins une dose ne dépasse 35 %, selon les chiffres de Santé publique France. La Guyane serait même le département le moins vacciné de France. C'est d'autant plus inquiétant que les outre-mer ont des prévalences de diabète, d'obésité et d'autres comorbidités avérées à la covid-19 bien supérieures à l'Hexagone. Pire, alors que les Antilles et la Guyane ont connu et la Guyane ont connu une quatrième vague particulièrement sévère et meurtrière, aucun sursaut vaccinal ne semble survenir. Nous cherchons tous à comprendre les raisons de cette réticence vaccinale, et la mission présidée par Bernard Jomier y consacre ses travaux en ce moment. Sont évoqués, tour à tour, la défiance envers le gouvernement central, la sensibilité à toute une série de, le traumatisme

l'agence régionale de santé organise des opérations de « vaccinobus » dans les différentes communes de l'île. Des opérations de vaccination éphémères sont également organisées dans des maisons de quartier ou des salles des fêtes.

de nombreuses opérations de vaccination éphémères ont été lancées, notamment dans certains atolls reculés. Il faut rester ingénieux, souple et inventif pour essayer d'élargir au maximum cette couverture vaccinale, dont vous avez relevé qu'elle était encore largement insuffisante dans certains territoires.

je n'évoque malheureusement pas les taux de vaccination contre le covid-19 de la population antillaise, mais le taux de contamination de celle-ci au chlordécone. Pendant deux décennies, la France a continué à autoriser un produit dont la toxicité était avérée. Elle a laissé les cultivateurs de bananes s'empoisonner et tout empoisonner autour d'eux, et ce pour plusieurs siècles, car nous sommes incapables de décontaminer les sols et les réserves d'eau. ans plus tard, le rôle de l'État dans ce scandale sanitaire hors norme, étayé en 2019 par une commission d'enquête parlementaire, n'est reconnu que du bout des lèvres. La reconnaissance du lien de causalité entre le chlordécone et le cancer de la prostate n'est toujours pas établie par les autorités françaises. Les victimes n'ont jamais été indemnisées et votre quatrième plan chlordécone, présenté en mars, ignore largement ces enjeux. Quel rapport avec le sujet qui nous occupe, me demanderez-vous ? Je le crois pourtant évident. Si la Guadeloupe et la Martinique sont, et de très loin, les deux départements qui connaissent le plus faible taux de vaccination- à peine à peine 35 % de la population a reçu au moins une dose, soit un taux beaucoup plus faible que tous les autres territoires d'outre-mer -, c'est bien sûr tout sauf un hasard, même si l'on peut évoquer d'autres raisons. La confiance envers la puissance publique, les autorités sanitaires, et même la science, est largement entamée, pour ne pas dire rompue.

fin 2018. Le Gouvernement est mobilisé pour que, face à cette pollution, l'État prenne sa part de responsabilité et avance sur le chemin de la réparation et des projets.

qui n'avaient jamais été tenues. Je pense par exemple à la reconnaissance du cancer de la prostate potentiellement causé par le chlordécone comme maladie professionnelle.

il n'y a aucun lit disponible au centre hospitalier de l'Ouest guyanais, en pédiatrie, à la maternité [ ...], aucun lit en service de médecine polyvalent, [ ...] et surtout aucun lit en réanimation ». Ce cri de détresse de Crépin Kezza, chef des urgences de ce centre, montre le décalage entre la métropole et nos collectivités d'outre-mer. les disparités sont importantes, nous souhaitons néanmoins interroger le Gouvernement sur ce décalage. Décalage dans le temps, décalage dans l'intensité, la vague d'épidémie qui frappe qui frappe quasiment l'ensemble de nos collectivités d'outre-mer depuis l'été est un véritable choc et nous ne pouvons que soutenir nos concitoyennes et concitoyens ultramarins. La Nouvelle-Calédonie, jusqu'à présent, accuse plus de 100 morts en un mois sur ses 280 000 habitants. En Guadeloupe, où la situation s'améliore, ce taux demeure supérieur au seuil d'alerte. Nous nous entendons tous pour dire que la campagne vaccinale permet de renverser ces tendances dramatiques. Mais cela ne suffit pas. Le manque de lits, le tri des patients, les personnels épuisés sont le résultat de sous-investissements chroniques. À Mayotte, on compte 300 lits au CHU alors qu'il en faut 900 en temps normal pour couvrir les besoins. En Guyane, on décompte 55 généralistes pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale est de 104. Ces déserts médicaux sont dénoncés chaque année, mais aucun véritable plan de rattrapage n'a été mis en place pour y remédier. Ces mêmes populations, qui souffrent là d'habitat insalubre, ici de coupures d'eau quotidiennes, ont une histoire bien à elles, qui alimente une crainte face aux injonctions du pouvoir éloigné d'elles, à Paris.

notamment, j'y reviendrai, à travers le Ségur de la santé, qui s'attaque à un certain nombre de problèmes structurels que vous soulevez.

je m'en tiendrai à quelques faits marquants : 53 000, c'est le nombre de personnels qui ont déjà été revalorisés, en cumulé, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et en Guyane ; 1,57 milliard d'euros, c'est le montant du plan

des actions très concrètes, qui concernent nos concitoyens et les professionnels de santé. Je citerai par exemple en Guadeloupe un projet d'investissement médico-social de plusieurs millions d'euros pour rénover les bâtiments ; en Martinique, le développement d'une plateforme numérique en mode SaaS,, qui va permettre aux patients d'accéder à une information rapide au sujet

je tiens à associer mon collègue Gérard Poadja, sénateur de la Nouvelle-Calédonie, à ma question. Il y a à peine un an, la Nouvelle-Calédonie tenait une deuxième consultation sur son autodétermination. Après une mobilisation historique, le « non » l'emporte, conduisant les indépendantistes à solliciter une troisième consultation, dont la date a été fixée par le Gouvernement au 12 décembre prochain. Toutefois, dans un contexte sanitaire inquiétant, des voix - majoritairement indépendantistes - se sont élevées pour envisager le report d'un tel référendum, par crainte d'une forte abstention. Face à un taux d'incidence élevé, à un taux de vaccination de 42 % insuffisant, et à des capacités d'accueil hospitalières en surchauffe, et après le décès de 160 de nos compatriotes calédoniens, le Gouvernement et le haut-commissaire ont acté la prolongation du confinement pour deux semaines. Monsieur le secrétaire d'État, malgré les renforts de près de 300 soignants volontaires de la réserve sanitaire, et alors que le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu, est actuellement sur place pour faire le point sur l'évolution de la pandémie, craignez-vous que les conditions sanitaires ne permettent pas la tenue de ce troisième référendum ? Quel dialogue envisagez-vous avec l'ensemble des parties prenantes à cet égard ? La parole

Nous devons être prêts pour le 12 décembre, date arrêtée en juin après des discussions approfondies avec toutes les composantes politiques calédoniennes.

Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 31 cas de covid identifiés depuis le début de la crise - 31 cas guéris -, mais c'est aussi 90 % de la population vaccinée en première dose - un taux sinon satisfaisant, du moins exemplaire -, et 88 % de la population vaccinée en seconde dose. Peut-être d'ailleurs Saint-Pierre-et-Miquelon aurait-il pu servir de modèle, à bien des égards, s'agissant de la territorialisation des mesures appliquées aux territoires ultramarins, voire hexagonaux. Depuis le 4 octobre ont été mises en place de nouvelles conditions de circulation, de et vers les outre-mer depuis l'Hexagone.

Comment justifier auprès d'une population presque intégralement vaccinée que les tests PCR ne seront pas remboursés, alors qu'ils sont imposés par la puissance publique ? Il ne s'agit pas de tests de confort, si tant est que le Gouvernement entende les maintenir.

canadienne prévoit bien un test. Le communiqué de presse précise qu'il doit s'agir d'un test PCR, compte tenu du fait que le Canada n'accepte pas les tests antigéniques. J'invite évidemment toutes celles et tous ceux qui se rendent à Saint-Pierre

là aussi à clarifier les choses : pour les personnes vaccinées qui seraient toutefois invitées à réaliser un test PCR, celui-ci sera bien pris en charge par l'assurance maladie.

Mme Viviane Artigalas. Monsieur le secrétaire d'État, alors que la France métropolitaine s'inscrit dans le plan de relance et réfléchit à la « France de demain », les départements et territoires d'outre-mer sont toujours en situation de gestion de crise. La situation de leurs entreprises est rendue extrêmement compliquée par l'état d'urgence sanitaire. La persistance des mesures de restriction a entraîné l'arrêt de nombreux secteurs essentiels à leur économie, à commencer par le tourisme, dans des proportions sans commune mesure avec ce qu'a subi la métropole. De plus, les entreprises sont très affectées par les difficultés d'approvisionnement. Elles subissent une hausse du prix du fret et des matières premières. Cela est d'autant plus délétère pour l'économie ultramarine que son marché est de taille plus réduite. Pour les entreprises qui souhaitent se pérenniser et celles qui viennent à peine de se créer, ce contexte compromet gravement leur viabilité et constitue une menace pour l'emploi. Malgré les annonces du Gouvernement concernant les nouvelles modalités d'accompagnement de l'État, les milieux économiques jugent certaines propositions insuffisantes, inadaptées ou imprécises. Monsieur le secrétaire d'État, que comptez-vous faire pour adapter les conditions d'éligibilité au fonds de solidarité au contexte ultramarin, dont le tissu d'entreprises est essentiellement fait de très petites entreprises pour accélérer le traitement des dossiers et le rendre plus souple pour les entreprises ? Comptez-vous prolonger le dispositif d'aides jusqu'au 31 décembre 2021, en particulier pour le secteur touristique, qui a vu sa saison réduite, et accuse donc une lourde perte de chiffre d'affaires ?

particuliers, le déploiement des divers dispositifs a été, je crois, rapide et efficace, et souligné par tous. La mise en oeuvre de l'activité partielle, par exemple, a permis de soutenir les ménages. Le suivi des besoins précis des populations, notamment des plus précaires, a été attentif ; il a donné lieu, quand c'était nécessaire, à des appuis plus ciblés encore.

L'impact sur l'emploi global est resté limité en raison du secteur public dans ces territoires. Le choc de la crise a été contrasté selon les géographies. En 2020, le PIB a ainsi reculé de 4,2 % à La Réunion et de 3 % aux Antilles. Le repli est estimé autour de 6 % en Nouvelle-Calédonie et à 7,6 % en Polynésie, soit une évolution similaire d'ailleurs à celle de la France hexagonale, où le repli a été de 7,9 %.

Nous sommes de nouveau dans une situation qui appelle un traitement différencié outre-mer. Vous avez raison sur ce point et nous partageons cette analyse avec les acteurs économiques, avec qui nous sommes naturellement en relation régulière. Leurs propositions sont prises en compte. La trajectoire d'extinction du fonds de solidarité a ainsi été stoppée pour les territoires qui, au mois d'août, ont été soumis à l'état d'urgence sanitaire et placés sous le régime du confinement ou du couvre-feu pendant au moins vingt jours. Vous voyez, madame la sénatrice, nous nous évertuons à rester pragmatiques, au plus près des situations locales, pour plus d'efficacité.

il n'en est pas moins vrai que des difficultés demeurent. Lors de la séance des questions au Gouvernement du 22 septembre dernier, j'ai eu à faire remonter les plus urgentes. La prise en compte par l'État d'une demande de financement d'un laboratoire d'analyse intra-muros à l'hôpital nous satisfait et nous vous en remercions. Cependant, l'autre grande urgence pour la population saint-martinoise est bien la prise en charge des évacuations sanitaires. Il existe une réelle perte de chance pour les Saint-Martinois du fait que nous ne pouvons pas bénéficier de l'hélicoptère de la sécurité civile de la Guadeloupe, et que le décollage des avions n'est pas possible de nuit. Je reste persuadée- et je ne suis pas la seule -qu'un troisième hélicoptère dans la grande zone Antilles, dédié aux îles du Nord et mutualisé entre les deux hôpitaux, la gendarmerie, la sécurité civile, les sauveteurs en mer, seule solution pérenne qui permettrait de garantir à la population saint-martinoise une prise en charge répondant aux mêmes exigences que celles qui sont requises sur le territoire hexagonal en termes d'accès aux soins. J'espère, monsieur le secrétaire d'État, que cette solution est à l'étude ... Par ailleurs, la gestion de la crise sanitaire à Saint-Martin, en particulier l'instauration d'un passe sanitaire, mériterait des ajustements. La double insularité et le partage de l'île rendent cette gestion compliquée. La fragilité économique et sociale se verrait aggravée par la mise en place d'un passe sanitaire sans ajustement. Économiquement, nous serions concurrencés par le côté néerlandais, dont nous n'avons pas la maîtrise : ce qui est interdit en France ne l'est pas de l'autre côté de l'île.

évidemment, comme tant d'autres, à de nombreux enjeux depuis le début de la crise sanitaire. Cette crise a révélé, amplifié parfois, un certain nombre de difficultés préexistantes. Cet hôpital est membre du groupement hospitalier territorial (GHT) des îles du Nord, lequel place sous direction commune les centres hospitaliers des deux îles, ainsi que les deux Ehpad. L'hôpital de Saint-Martin fonctionne ainsi en partenariat avec un laboratoire et un cabinet de radiologie

en Guadeloupe. Cela m'amène à la question des évacuations sanitaires, à la particularité de ce centre hospitalier et à la charge très lourde des évacuations sanitaires vers la Guadeloupe et la Martinique. Un marché existe, dont le budget annuel est d'environ 2,5 millions d'euros. Le ministère des solidarités et de la santé a pris en compte cette charge et un financement complémentaire est en cours de déploiement. La question d'un hélicoptère supplémentaire dans la zone est posée, car le décollage et l'atterrissage de nuit sont très problématiques. Un audit devrait être demandé conjointement par l'agence régionale de santé et la préfecture à ce sujet.

d'application entre les parties néerlandaise et française de l'île, nous avons bien conscience des interrogations que cela peut soulever sur le terrain. Pour autant, je pense que nous aurions tort de nous comparer avec la partie néerlandaise, qui n'a donc pas mis en place

Les sénateurs de l'Union Centriste estiment que la politique de vaccination devrait prendre en compte les facteurs socioculturels freinant la campagne de vaccination, les raisons historiques et humaines à l'origine de la défiance de la population vis-à-vis du Gouvernement.

En outre, il convient de prendre en considération la résistance sociale des Ultramarins, qui n'ont malheureusement pas conscience de l'urgence de la situation. La communication est souvent contradictoire et, assurément, votre moyen d'action pour infléchir la courbe de l'épidémie, c'est la pédagogie. Il faut comprendre à qui l'on s'adresse. La méfiance envers les médias et l'importance accordée à la médecine traditionnelle sont autant de freins à la progression de la vaccination. Aux Antilles, les gens sont habitués à se soigner par des plantes, avec des sirops à base d'herbes à pic, qu'ils estiment suffisants pour renforcer l'immunité contre la covid. Pourtant, ce traitement complémentaire n'est pas un traitement alternatif. N'oublions pas non plus le poids de l'Histoire. Plusieurs de nos collègues ont rappelé le scandale du chlordécone, ce pesticide nocif massivement utilisé aux Antilles jusque dans les années 1990, alors qu'il était interdit dans l'Hexagone. Ces circonstances permettent parfois de comprendre pourquoi l'État n'est plus considéré comme légitime, ou encore pas assez protecteur, aux yeux d'une partie de la population. Cette posture de résistance face aux décisions du Gouvernement est souvent mal comprise. Comment comptez-vous, monsieur le secrétaire d'État, agir pour débloquer la situation et augmenter le taux de couverture vaccinale outre-mer ? Comment entendez-vous relever le défi de la communication ? Quel est le rôle des influenceurs et des personnalités politiques pour faire passer les messages à

je la rappelle : en continuant à compter sur la très forte mobilisation de l'ensemble des autorités sanitaires et des professionnels de santé ; en vainquant les réticences persistantes contre la vaccination la démultiplication des campagnes de communication et en luttant contre les. Cela passe également par des déclarations de responsables politiques,

reste importante. Il y a probablement dans les territoires, dans une approche plus communautaire, des relais d'opinion que nous devons probablement mobiliser davantage afin de convaincre la population de se faire vacciner, de renouer avec la confiance dans la raison, dans la science, dans la vaccination.

d'État, alors que les premières vagues nous ont plus ou moins épargnés, cette quatrième vague a été meurtrière et a révélé les limites des moyens existants, tant humains que matériels. À ces carences se sont ajoutées des difficultés liées à une très mauvaise communication de la part de la directrice générale de l'ARS, qui n'a pas facilité les relations avec la population et même avec certains médias. La mise en place tardive des restrictions concernant les vols transatlantiques n'a pas permis d'éviter cette vague et les propos irrespectueux, moralisateurs et méprisants, notamment sur les médias nationaux, qui ont relayé certaines ont compliqué, dans un contexte de méfiance,

certaines conséquences de la propagation du variant delta ont été amplifiées en raison des retards structurels que connaissent nos territoires en matière de santé. Des professionnels venus en renfort ont constaté les manques

Comme je l'ai souvent rappelé dans cet hémicycle, en particulier à chaque discussion budgétaire, nos établissements de santé, qui sont déjà largement sous-dotés, doivent en outre faire face à des surcoûts importants liés au fonctionnement, à la maintenance et à l'amélioration continue de la qualité. Il faut souligner l'implication des élus locaux au sein du comité de suivi présidé par le préfet. Malheureusement, les médecins de ville n'ont pas été suffisamment pris en compte.

le GIP en un DAC, un dispositif d'appui à la coordination. Je rappelle d'ailleurs que la mise en place d'un DAC est une obligation légale depuis 2019.

Mme Micheline Jacques. Monsieur le secrétaire d'État, chaque fermeture des frontières équivaut à mettre Saint-Barthélemy à l'arrêt. Pour sortir de ce fonctionnement sur courant alternatif, une des clefs est la réduction de la dépendance à l'extérieur en matière d'offre de soins. La gestion de l'épidémie a montré, s'il en était besoin, que l'adaptation à la réalité de l'île a été gage d'efficacité et l'implication de la collectivité a sans nul doute permis d'optimiser les dispositifs de gestion de crise. Dès le premier confinement, elle a pris l'initiative d'équiper massivement l'île en capacités de tests PCR rapides. Un protocole de test et des décisions concertées ont permis de juguler les pics de contamination avec des mesures de restriction relativement limitées. Le pragmatisme commande désormais de pérenniser et de formaliser cette implication- c'est du reste ce que souhaite la collectivité de Saint-Barthélemy depuis plusieurs années -pour disposer d'une organisation et d'une offre de soins davantage territorialisées. La gestion du service de proximité de la sécurité sociale favorisera l'amélioration du service aux usagers. Il s'agit de plus d'exploiter les possibilités offertes par le statut d'hôpital de proximité pour aller vers plus d'autonomie, en réduisant le nombre d'échelons décisionnels, tout en étoffant l'offre de soins. Ce dernier objectif suppose des moyens matériels et de sécurisation des évacuations sanitaires qui doivent être pensés à l'échelle du groupement hospitalier formé avec Saint-Martin.

de dresser un état des lieux précis et de mettre sur la table toutes les solutions possibles pour repenser une offre de soins étoffée à Saint-Barthélemy. Cet amendement a été soutenu par le ministre des outre-mer. Pouvez-vous me confirmer, monsieur le secrétaire d'État, que le ministre des solidarités et de la santé y est également favorable ?

professionnels de santé qui exercent en Ehpad ont suivi un schéma vaccinal complet. Il faut continuer la pédagogie et expliquer aux professionnels de santé l'impérieuse nécessité de se faire vacciner.

elle l'est tout particulièrement dans la collectivité de Guyane, où le taux d'incidence est désormais le plus élevé- plus de 500 cas pour 100 000 habitants -et où les taux de vaccination restent très bas, avec seulement 30 % des douze ans et plus ayant reçu les deux doses. Les mesures de freinage ont encore été renforcées jeudi dernier avec la fermeture de nombreuses classes. À titre personnel, et comme vous le savez, j'ai pris mes responsabilités et appelé sans détour à la vaccination. Je persiste à défendre cette ligne, en appelant sans réserve mes concitoyens à se protéger et à protéger les autres. La dégradation rapide de la situation dans nos outre-mer a conduit, fin août, la mission commune d'information du Sénat destinée à évaluer les effets des à orienter ses travaux sur l'évaluation de la gestion de la crise par le Gouvernement dans les territoires ultramarins. Cette prise en compte s'est faite à la demande du président du Sénat, Gérard Larcher, et à la suite d'échanges avec les collègues qui alertaient sur la situation inédite dans leurs territoires. Saluant cette décision, j'ai proposé que les sénateurs ultramarins soient associés à ce travail afin que soit portée la voix des outre-mer par ceux qui en sont les représentants. Une première audition générale s'est ainsi tenue il y a une semaine, en commun avec les membres de la délégation sénatoriale aux outre-mer. Des tables rondes géographiques suivront pour apprécier la situation dans chacun des territoires. Je formule le voeu que cette mission avance des recommandations tant sur le plan sanitaire que sur les plans économique et social afin de répondre à l'urgence actuelle, mais aussi de tirer des leçons de long terme sur l'offre de soins en outre-mer. Après les nombreux échanges que nous avons eus ce soir, je voudrais retenir deux enseignements : l'un sur la solidarité nationale, qui s'est notamment manifestée à travers les prouesses qui ont été réalisées en matière d'évacuation sanitaire ; l'autre sur notre capacité à préparer « l'après », c'est-à-dire à anticiper une probable nouvelle vague et à reconstruire à la suite des dégâts multiples causés par cette pandémie, qu'ils soient humains, économiques, sociaux ou psychologiques. Au nom de la solidarité nationale, des moyens exceptionnels ont été déployés pour contrer la quatrième vague. Au total, plus de 2 800 soignants ont été envoyés en renfort dans nos différents territoires et nous saluons avec reconnaissance leur engagement. De nombreuses évacuations sanitaires ont été organisées. Grâce à l'opération Hippocampe, un pont aérien entre les Antilles et Paris s'est mis en place, permettant l'évacuation de 48 patients chaque semaine. Une première mondiale a même eu lieu : le 18 septembre, 8 patients en réanimation ont été évacués par avion de la Polynésie vers l'Hexagone, alors que 16 000 kilomètres séparent Papeete de Paris. Jamais un transport de malades d'une telle ampleur et à pareille distance n'avait été réalisé. À l'image des TGV médicalisés mis en place dans l'Hexagone pour soulager les hôpitaux proches de la saturation, une prouesse technique a été réalisée avec la transformation d'un avion de ligne en service de réanimation. La crise a rendu possible ce qui paraissait, il y a encore quelques semaines, presque impossible. C'est une leçon à retenir. Mais nos territoires ne pourront pas compter uniquement sur les évacuations sanitaires, si utiles soient-elles, pour faire face aux vagues épidémiques. Au terme de ce débat, il nous faut également tirer des enseignements pour mieux préparer nos territoires aux autres crises sanitaires, malheureusement prévisibles. Je conclurai par deux observations. Tout d'abord, vous l'avez dit, les uns et les autres, plusieurs facteurs peuvent expliquer l'ampleur de la crise en outre-mer : bien sûr de faibles taux de vaccination, mais aussi des taux de comorbidité plus importants, l'éloignement de l'Hexagone qui rend les évacuations, malgré les prouesses récentes, plus difficiles des habitats insalubres encore trop nombreux sur certains territoires, qui empêchent la bonne application des mesures de confinement. Toutes ces explications sont recevables, mais on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion en profondeur sur l'offre de soins en outre-mer. Mme Cécile Courrèges, inspectrice générale des affaires sociales, indiquait d'ailleurs, lors de son audition par la mission commune d'information : s'agissant des Antilles : « Il ne faut pas revenir au même niveau de soins critiques qu'avant la crise, il faut un niveau plancher supérieur pour avoir une capacité de rebond un peu meilleure qu'avant la quatrième vague. » De façon plus générale, je souhaite aussi rappeler que, selon une étude de la direction trois territoires ultramarins arrivent en tête des régions les plus touchées par la désertification médicale. Ainsi, 44 % des Guyanais et 18 % des Martiniquais et des Guadeloupéens vivent dans des zones sous-denses, c'est-à-dire avec un accès à moins de 2,5 consultations par an et par habitant. On constate des pénuries de professionnels libéraux et la Cour des comptes notait, dans un rapport de 2014, que de nombreuses évacuations sanitaires sont aussi le fait de l'absence de certaines spécialités dans les territoires. Si les moyens exceptionnels déployés sont strictement la réponse à une crise brutale et inédite, ils ne seront pas appelés à durer. Il n'en est pas de même, s'il s'avère que ces moyens sont venus compenser des fragilités structurelles du système de soins en outre-mer. Sur tous ces sujets, notamment sur le dimensionnement de l'offre médicale, il appartiendra à la mission commune d'information d'apporter des éléments de réponse et d'éclairage et je félicite encore son président, Bernard Jomier, et ses deux rapporteurs, Jean-Michel Arnaud et Roger Karoutchi, pour leur implication. Ce travail difficile, mais nécessaire, doit conduire à une meilleure autonomie et à une plus grande résilience sanitaires de nos territoires. Je suis convaincu que la délégation sénatoriale aux outre-mer, à laquelle j'appartiens et qui a souhaité le débat de ce soir- je remercie son président, Stéphane Artano, et tous nos collègues qui sont intervenus avec force et émotion apportera sa pierre à ce travail fondamental. Il nous faut pouvoir tirer les leçons des événements récents et surtout bâtir des solutions pérennes. Nous en